La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, a demandé de compléter l'ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 25 octobre 2018 par un débat portant sur le thème de « la scolarisation des enfants en situation de handicap ». Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 16, alinéa 2, du règlement, la proposition de création de trois commissions spéciales chargées d'examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission. Je soumets donc cette proposition au Sénat. Il n'y a pas d'opposition Il en est ainsi décidé. Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des trente-sept membres de chacune de ces commissions spéciales aura lieu en séance publique, demain, à

elles-mêmes ou faire appel à tout mandataire de leur choix, qu'il s'agisse de leur conjoint, d'un concubin, d'un huissier de justice, d'un fondé de pouvoir. La commission des lois du Sénat a entendu donner valeur législative au principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce. cela ne me paraît pas respecter ce qui relève du domaine du règlement. De telles dispositions sont en effet antérieures à la loi de 1971, qui donne aux avocats un monopole d'assistance et de représentation en justice. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dérogations au monopole de représentation par avocat antérieures à la loi de 1971 ont vocation à rester réglementaires. Je souhaite donc que ces dispositions puissent demeurer de nature réglementaire.

adoptée par la commission des lois. Dans le droit actuel, les parties peuvent non seulement se défendre elles-mêmes, mais aussi se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce. Ce principe est défini par l'article 853 du code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'une dérogation manifeste au principe de représentation obligatoire par avocat prévu à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

exception pour les caisses de sécurité sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l'aide sociale et le contentieux technique. Les personnes handicapées, malades, accidentées ou invalides devront en revanche être représentées par un avocat pour faire reconnaître leurs droits. Cette mesure pénaliserait indéniablement des publics qui, en raison de leur situation, ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour engager des contentieux. S'ajoute à cela qu'aucune mesure ne prévoit la prise en charge du coût du recours à un avocat. La représentation obligatoire pour ces contentieux en appel conduirait aussi à exclure des associations qui, comme la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, oeuvrent pour l'accès au droit des personnes fragilisées, en leur apportant la technicité et l'appui qu'implique la complexité des procédures juridiques. Cet amendement vise à créer un « défenseur social ». Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés.

précité énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la cour d'appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial. Dans la mesure où des dérogations existent déjà dans le projet de loi, nous souhaitons voir renforcé l'accès au droit. Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés. Notre

que l'organisation judiciaire en cette matière va être profondément revue au 1 janvier 2019, puisque des pôles sociaux seront créés dans les tribunaux de grande instance, en lieu et place des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des commissions départementales d'aide sociale. Il pourra être fait appel des décisions rendues par le TGI en ces matières devant une cour d'appel spécialement désignée. Le projet de loi étend la représentation obligatoire par avocat à ces contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, mais seulement en appel. La problématique n'est pas la même en appel qu'en première instance. En effet, dès lors qu'une partie aura pu se défendre librement en première instance, et ce sera le cas en matière sociale, mais qu'elle n'aura pas eu gain de cause, il me paraît opportun et rationnel qu'elle soit tenue de constituer avocat en appel pour assurer une meilleure représentation de ses causes. Je m'inscris d'ailleurs dans la continuité de ce que le Sénat avait adopté dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXI siècle. Je précise en outre que le dispositif proposé dans cet amendement ne me semble pas pas correspondre à son objet, car son adoption reviendrait à permettre aux organismes de sécurité sociale d'être défendus en appel, outre par un avocat, par un défenseur social. Or les auteurs de l'amendement doivent sans doute viser toutes les parties au litige. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable

en appel et devant la cour d'appel spécialement désignée pour les litiges qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Cette extension se justifie par la complexité de la matière, pour laquelle l'intervention d'un spécialiste du droit nous semble bénéfique pour le justiciable en raison du conseil juridique qui lui est apporté. Je n'ignore évidemment pas le rôle qu'assurent actuellement les associations de personnes handicapées, accidentées, malades ou invalides, qui pourront bien entendu continuer à exercer leurs missions de conseil et de soutien. Néanmoins, la possibilité de représentation des parties par un défenseur social ne répond pas à l'objectif de protection du justiciable dans le cadre d'une instance d'appel, qui doit être concentrée, je le rappelle, sur les questions de droit. de droit. Ces dernières supposent suffisamment d'expertise pour justifier la présence d'un avocat. De même, devant la cour qui connaît en premier et dernier ressort du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et qui oppose exclusivement les employeurs aux caisses, l'intervention d'un défenseur social me semble sans objet. L'objectif est pour nous d'étendre avec discernement le périmètre de la représentation par avocat et non de créer une nouvelle dérogation. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable

d'où je viens, mais la qualité de ces associations, sur le plan technique, à propos de questions juridiques très complexes et particulières, est souvent bien meilleure

s'agissant des actes de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation, ainsi que des actes de notoriété suppléant les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par la suite d'un sinistre ou de faits de guerre. La commission a estimé qu'un tel transfert s'inscrivait dans une logique d'uniformisation des règles de compétence applicables à la délivrance des actes de notoriété. En effet, le code civil prévoit deux autres hypothèses dans lesquelles

que les témoins qui comparaissent devant elle affirment qu'à leur connaissance personnelle tel fait est notoire. L'esprit du projet de loi de programmation pour la justice est, j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, de recentrer l'office du juge sur les tâches qui appellent incontestablement une intervention judiciaire et pour lesquelles le juge apporte une réelle plus-value, ce qui n'est pas le cas des actes de notoriété. Il s'agit également d'uniformiser les règles de compétence régissant les différents actes de notoriété établis établis dans diverses matières. En effet, le code civil prévoit déjà quatre autres dispositions relatives à des actes de notoriété tous dressés par des notaires : les actes de notoriété dressés pour la constitution du dossier de mariage, en matière successorale, en matière d'indivision, ainsi qu'en matière de prescription acquisitive immobilière. Je n'ignore pas la question du coût de la délivrance d'un tel acte, que vous avez relevée. Je souligne toutefois que ce coût sera limité, puisque les émoluments des notaires sont réglementés. En l'occurrence, l'émolument fixe s'élèvera à 57,69 euros. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que le nombre de ces actes de notoriété se limite à une dizaine par an. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

en l'espèce, celle-ci se fait en faveur d'acteurs privés et emporte un coût pour l'usager et une forme d'appropriation lucrative du service public. Nous nous opposons donc à ce qui apparaît comme le moyen par lequel on rend payant un service aujourd'hui gratuit, ce qui va peser nécessairement sur les plus vulnérables et peut-être leur interdire le recours à certains services ou l'exercice de certains droits. Par cet amendement n° 126, nous nous opposons

En matière de filiation, la déjudiciarisation de l'acte de notoriété s'inscrit déjà dans la continuité de missions actuelles confiées aux notaires, lesquels sont aujourd'hui compétents pour les actes de reconnaissance en matière de filiation. Par ailleurs, cette déjudiciarisation de filiation. Par ailleurs, cette déjudiciarisation s'opère au bénéfice des notaires et il faut ici les considérer comme des officiers publics et ministériels,

devant faire face à un problème médical d'infertilité et qui a le choix entre le notaire ou le juge pour donner son consentement. Cette intervention du notaire est adaptée, car il s'agit d'informer le couple sur les règles de filiation dérogatoires qui s'appliquent dans le cadre de l'AMP avec tiers donneur. L'intervention du juge, en revanche, ne se justifie pas : il n'exerce là aucune fonction juridictionnelle, se contentant de recueillir un consentement. La modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est donc une mesure d'administration de la justice, qui s'inscrit dans la démarche globale de simplification des procédures qui anime ce projet de loi. Confier ainsi exclusivement le recueil du consentement au seul notaire ne pose aucune question éthique et a donc davantage sa place dans le projet de loi de programmation pour la justice

la commission. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois de bioéthique, il n'était pas selon nous pertinent de les

Nous contestons ce nouveau dispositif, non seulement injuste, mais également de nature à créer une certaine confusion chez le justiciable. Injuste, car, dans le droit positif, les décisions de révision des pensions sont le fait du contentieux judiciaire, plus précisément du juge aux affaires familiales. Le dispositif actuellement en vigueur, bien qu'imparfait, permet l'évaluation des situations par le juge par un réexamen sur le fond des situations sociales et financières des deux parents, ainsi que des besoins de l'enfant, on parvient à faire respecter au mieux l'intérêt supérieur de celui-ci. Avec la déjudiciarisation des révisions des pensions proposée par le Gouvernement, on entre dans l'ère de la non-individualisation des décisions confiées à un organe administratif, qui ne présente pas les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance que le juge aux affaires familiales. On peut craindre que les révisions ne fassent désormais l'objet d'une barémisation. Enfin, comment expliquer rationnellement que le juge aux affaires familiales sera toujours compétent en matière de fixation des droits de visite, de placement des enfants et de leur hébergement lorsqu'il sera destitué des contentieux ayant trait à la pension alimentaire ? Alors que le Gouvernement se targue de procéder à une simplification de notre système judiciaire, tel dispositif va à l'encontre de cet objectif, en le complexifiant par un procédé inique pour les familles les plus instables et précaires. Pour cette raison, nous demandons la suppression de l'article 6. Quel ? Cet amendement vise à supprimer l'article 6, relatif à l'expérimentation de la révision des pensions alimentaires par les caisses d'allocations familiales,

d'une part, sur le barème déjà utilisé par les juridictions et les avocats, ce qui sera source d'une meilleure prévisibilité pour les parents et, d'autre part, sur les documents échangés contradictoirement par les parents.

d'une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée par le juge en fonction d'une situation donnée- besoins des enfants, revenus du père et de la mère. cette situation évolue, un nouveau débat judiciaire doit s'ouvrir entre les parties. Si les parties sont d'accord et concluent une convention,

Mme Éliane Assassi. L'article 6 consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette déjudiciarisation est plus qu'inquiétante, puisqu'elle aboutit à une atteinte d'une exceptionnelle gravité

présentation, madame la ministre, pour vous faire part de l'avis des membres du barreau de Paris sur cet aspect de votre projet de loi : « C'est une atteinte grave à la démocratie et au principe de la séparation des pouvoirs. Dans un État de droit, il est impossible qu'une décision définitive d'un juge judiciaire soit modifiée par le directeur d'une CAF. Cela se ferait nécessairement au détriment des Français les moins riches, car les CAF ne connaissent pas l'intégralité des revenus des plus aisés, qu'ils proviennent de l'étranger ou des capitaux, notamment. Cette réforme créerait une inégalité entre les Français, alors que la pension alimentaire constitue un élément essentiel de l'équilibre d'un divorce. Il est intolérable

commission ? Cet amendement prévoit une décision du juge aux affaires familiales pour autoriser les caisses d'allocations familiales à réviser les pensions alimentaires.

depuis le 1 avril 2018, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut déjà donner force exécutoire à l'accord par lequel les parents qui se séparent fixent le montant de cette contribution, sous certaines conditions. L'expérimentation, pour être utile, doit donc viser d'autres hypothèses que celle de l'accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire. Afin de permettre une

qui ne produirait pas les renseignements nécessaires pour apprécier la demande, l'organisme saisi pourrait appliquer un forfait pour le montant de la pension. Ce dispositif est donc incitatif pour les parents ; il permettra de délivrer dans des délais brefs un titre exécutoire établi en fonction de documents qui seront échangés contradictoirement, sur le fondement d'un barème connu et objectif.

après une fixation initiale par le juge ou par accord entre les parents, en dehors de toute question relative à l'autorité parentale. J'entends également que certains craignent une sorte de conflit d'intérêts pour les organismes désignés. Ils soutiennent en particulier que les CAF seraient juge et partie, puisqu'elles distribuent des prestations familiales en cas de carence ou d'insuffisance de la pension alimentaire. Elles pourraient donc être tentées d'en augmenter le montant pour payer moins de prestations. En premier lieu, comme toute personne morale chargée d'une mission de service public, la CAF, dans son fonctionnement, répond aux exigences de neutralité et d'impartialité- il est important de le souligner. Il lui appartient, le cas échéant, d'adapter son organisation interne en conséquence. En deuxième lieu,

en troisième lieu, la CAF n'aurait aucun intérêt à majorer sans justification le montant des pensions alimentaires. Cela entraînerait presque automatiquement la défaillance du débiteur et la CAF serait alors obligée de verser la prestation compensatoire correspondante. En outre, dans ces situations, la CAF doit lancer une procédure de recouvrement qui conduit à un travail supplémentaire, coûteux et inutile pour elle. Cette expérimentation que je propose apparaît donc mesurée Elle devrait permettre, par une meilleure prévisibilité du montant de la pension, une relative pacification des relations entre les parents séparés.

restreindre le champ de cette expérimentation aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d'accord sur le nouveau montant de la pension. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de l'amendement,

pour l'instant intervenir qu'en matière de fixation ou de révision de pensions concernant des parents qui n'étaient pas mariés. Le nouveau dispositif permettrait d'intervenir cette fois pour réviser les pensions de tous les parents, qu'ils aient été mariés ou non. La commission a voulu en revanche écarter l'application de l'expérimentation en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l'application mathématique d'un barème, y compris lorsque l'un des parents n'a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le fait habituellement le juge. a également choisi de limiter les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l'article 6, dans sa rédaction initiale, donnait compétence aux caisses d'allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser lesquels, publics et ministériels, sans préciser lesquels, la commission a préféré confier cette compétence aux seules caisses d'allocations familiales, qui, comme le fait valoir le Gouvernement, interviennent déjà en la matière depuis le 1 avril 2018 et disposent par ailleurs d'un accès facilité aux informations nécessaires

2016 et appliqué depuis le mois d'avril dernier en cas d'accord entre les parties. Si votre objectif est effectivement de trouver un organisme public qui, en dehors de la justice, puisse modifier les pensions alimentaires en l'absence d'accord entre les parents, pourquoi ne proposez-vous pas aux services fiscaux de le faire ?

Mme la garde des sceaux. Cet amendement vise à simplifier le changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs, en supprimant l'intervention systématique du juge. Il s'agit là d'une simplification très importante, qui s'inscrit dans les objectifs de ce projet de loi. L'homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs

une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Les parents sont en effet les premiers garants de l'intérêt de leurs enfants et, bien souvent, la demande de changement de régime matrimonial intervient précisément pour

Pour les hypothèses résiduelles où il existerait un risque que l'un des parents ou les deux agissent en contradiction avec les intérêts de l'enfant mineur, un mécanisme de contrôle demeure prévu. Dans ce cas, si les intérêts des enfants ne paraissent pas respectés, le notaire, officier public et ministériel, tenu à un devoir renforcé d'information et de conseil, devra faire part de ses doutes aux époux. Il pourra ensuite, si la situation le justifie, saisir le juge des tutelles des mineurs, sur le fondement de l'article 387-3 du code civil. Dans ces situations, le contrôle judiciaire est prévu pour évaluer le changement envisagé. L'intervention judiciaire sera ainsi plus lisible et mieux comprise de la part de nos concitoyens, qui attendent cette simplification. Je souhaite donc que vous puissiez adopter cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs. Quel est l'avis de la commission ? J'ai peur de vous décevoir, madame la garde des sceaux ... Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité maintenir l'homologation par le juge des modifications du régime matrimonial en présence d'enfants mineurs. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, en 2015, le Sénat s'était déjà opposé à la suppression de cette homologation en présence d'enfants mineurs, estimant que l'intervention du juge permettait de vérifier que la modification est bien conforme à l'intérêt de la famille prise dans sa globalité, et pas seulement à celui des époux. La commission estime également inopportun de confier au notaire qui ne sera pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à la modification envisagée au nom de l'intérêt de leurs enfants le soin de saisir le juge, car cela le placerait dans une position délicate vis-à-vis de ses clients. En conséquence, l'avis est défavorable. La parole est

Benbassa, sur l'article. Le présent article vise à supprimer le contrôle du juge des tutelles pour certains actes concernant les majeurs protégés et à externaliser ce contrôle au profit des professionnels du chiffre et du droit. Encore une fois, nous assistons à la déjudiciarisation d'un domaine du droit parmi les plus importants pour la justice, celui du droit des majeurs protégés et du contrôle des mesures de protection judiciaire. Alors que les magistrats estiment que ce type d'actes ne représente pas une surcharge effective pour les juridictions, l'exécutif souhaite réaliser des économies en confiant le contrôle des comptes bancaires à des professionnels du chiffre et du droit. Cette mesure tend à éloigner le majeur protégé du contrôle du juge des tutelles, seul à même de protéger de manière impartiale et indépendante les majeurs sous protection judiciaire, alors que les abus tutélaires sont régulièrement dénoncés. Enfin, alors que la vérification des comptes par le directeur de greffe est aujourd'hui gratuite pour le majeur protégé, elle deviendrait payante en cas d'adoption du projet de loi et son coût serait mis à la charge de la personne protégée. Outre que, pour les professionnels du chiffre et du droit, l'ouverture de ce nouveau marché représente une manne de plus de 60 millions d'euros, cette disposition illustre la volonté du Gouvernement de faire peser le coût de la carence de l'État sur les justiciables les plus fragiles, ce qui est inadmissible. Il est clair que ce dispositif est proposé dans l'unique objectif de faire des économies. Une nouvelle fois, avec les dispositions de cet article, c'est l'accès à la justice des plus vulnérables qui est sciemment sacrifié.

dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il importe de renforcer la dignité des majeurs protégés dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il est essentiel de restaurer l'expression directe de leur volonté, chaque fois qu'elle est possible, et de supprimer les formalités qui apparaissent comme des obstacles illégitimes. À cette fin, je vous propose donc d'améliorer l'introduction de la procédure de protection judiciaire en imposant aux services qui saisissent le procureur de la République d'une demande de mise sous protection de motiver cette demande au regard d'une évaluation sociale et pécuniaire de l'intéressé. En effet, la saisine de l'autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise, qu'il s'agisse d'une perte d'autonomie, de l'isolement ou du refus des aides proposées, de décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou qui paraissent incohérentes, de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée, mais cette décision doit rester subsidiaire par rapport aux situations déjà en place. Le parquet ne peut assumer son rôle de filtre des demandes qu'au vu d'un état des lieux complet de la situation du majeur.

d'un PACS ou la décision de divorcer. Pour autant, la protection de la personne protégée reste assurée, puisque la personne en charge d'une mesure de protection devra être informée préalablement au dépôt du dossier en mairie, et elle bénéficiera d'un droit d'opposition au mariage plus large qu'aujourd'hui. En l'absence de la preuve de l'information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir, de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré. En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci, alors qu'il s'agit d'un divorce prononcé par un juge dans des conditions apaisées. Il est nécessaire d'ouvrir cette voie au majeur protégé qui souhaite divorcer sans l'obliger à passer par une phase contentieuse. L'acceptation du divorce relèvera alors de sa seule décision, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance. Dans la même ligne, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. Aujourd'hui, selon les médecins et les tuteurs, une autorisation du juge peut être sollicitée pour une extraction dentaire, même lorsque le majeur protégé et son tuteur sont d'accord pour suivre l'avis médical, ce qui retarde évidemment l'accès aux soins des plus vulnérables. par ordonnance est sollicitée pour poursuivre cette réflexion et mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles avec celles du code civil. Le contrôle du juge des tutelles sera également allégé pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant concernant l'administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur sous tutelle, ce qui correspond à la proposition n° 51 du rapport que m'a remis Mme l'avocate générale Anne Caron-Déglise, laquelle préconise de simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure et de supprimer nombre d'entre dès lors que ces opérations font l'objet d'un contrôle. Par ailleurs, l'article L. 5 du code électoral, qui permet au juge de supprimer le droit de vote des majeurs lorsqu'il prononce ou renouvelle une tutelle, est abrogé, ce qui représente une avancée très forte des droits des majeurs protégés. Le Président de la République avait annoncé, lors de son discours devant le Congrès à Versailles, le 9 juillet 2018, son souhait de voir les personnes sous tutelle

de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant les conditions des procurations pouvant être établies par des majeurs protégés et en interdisant ces procurations non seulement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais également aux personnes accueillant ou prenant en charge les majeurs sous tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. dispositif protecteur, ces personnes ne pourront pas non plus intervenir en tant que personnes assistantes au sens de l'article L. 64 du code électoral. Avec cette mesure, je vous propose réellement une très grande avancée pour les majeurs protégés

assez complet et qui touche beaucoup de sujets concernant les majeurs protégés. Vous proposez en partie la suppression du contrôle préalable du juge sur plusieurs décisions personnelles qui concernent les majeurs protégés.

curatelle de se marier ou de conclure un pacte civil de solidarité sans aucune autorisation du juge. Eu égard aux risques d'abus de faiblesse touchant des personnes vulnérables, il nous semble que l'intervention

alors qu'aujourd'hui le juge des tutelles décide au cas par cas. Là encore, une telle mesure ne nous semble pas opportune, car elle poserait de réelles difficultés, s'agissant notamment de personnes qui ne peuvent exprimer une volonté ou qui peuvent être influençables. Nous pensons qu'il faut faire confiance aux magistrats, qui apprécient chaque situation individuellement. Le droit en vigueur est d'ailleurs conforme à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, car il autorise les majeurs sous tutelle à voter dès lors que leur santé le leur permet. Par ailleurs, cela reviendrait à permettre aux majeurs sous tutelle d'être jurés d'assises, par exemple, puisqu'ils seraient inscrits sur les listes électorales, ce qui n'est sans doute pas tout à fait, j'imagine, l'objectif visé par le Gouvernement. En tout état de cause, ce sujet reste délicat et ne saurait être réglé à travers un simple amendement, sans que nous puissions aller plus loin. Le troisième point sur lequel nous sommes en désaccord, c'est l'allégement du contrôle du juge en cas d'acte médical grave sur la personne protégée. protégée. Dès lors que les situations d'urgence vitale sont dérogatoires, il nous semble qu'une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée requiert opportunément, là encore, le contrôle du magistrat. Autre sujet, l'ouverture du divorce accepté aux majeurs protégés nous semble moins contestable, disons les choses telles qu'elles sont, dès lors qu'ils seulement accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, tout en étant assistés ou représentés dans le reste de la procédure. Cela dit, la commission pense qu'elle manque d'éléments objectifs pour se prononcer véritablement sur cette mesure.

par Yves Détraigne et moi-même, concernant la suppression de l'autorisation du juge pour que le tuteur inclue certains frais de gestion dans le budget de la tutelle- recours à un avocat ou à un comptable, par exemple -ou conclue un contrat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers au nom de la personne protégée. Si le Gouvernement a supprimé la mention du conseil de famille en tenant compte, par ailleurs, de nos remarques, ce dont nous vous remercions, la suppression de tout contrôle de ces actes de gestion ne nous convainc pas.

je crois me souvenir que c'est le Sénat qui a ouvert pour la première fois la possibilité pour les incapables majeurs de voter dans les conditions qui sont actuellement prévues par le droit. C'est la Haute Assemblée qui était à l'origine, déjà, de cette avancée fondamentale. Pour autant, en l'espèce, par le biais d'un amendement,

va à l'encontre du principe de l'autonomie de la volonté de toutes les personnes qui peuvent s'exprimer. En matière de PACS, de mariage ou de divorce, le tuteur et le curateur continueront à intervenir pour protéger le majeur de tout abus sur son patrimoine. Il s'agit pour nous de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la réflexion de tous les acteurs qui ont participé au groupe de travail dont je me faisais l'écho à l'instant.

avec un accès limité au mécanisme des procurations. Pour toutes ces raisons, il me semblait important de pouvoir vous présenter ces dispositions, et, puisque vous êtes précurseurs en ces domaines, de pouvoir espérer un vote positif

dans la ligne de celles qui lui sont déjà confiées. Banquier du service public de la justice, la Caisse des dépôts et consignations dispose en effet de toutes les compétences utiles et mobilisables pour recevoir les fonds issus des saisies des rémunérations, pour les gérer et les répartir entre les créanciers. Il s'agit d'opérations de banque classiques, la seule particularité consistant, lors de l'opération de répartition, à déterminer la part qui revient à chaque créancier. Ce calcul procède de règles simples qui sont aisément automatisables. La CDC maîtrise en outre parfaitement les attributions qui lui sont transférées en matière d'expertise. Elle les pratique déjà pour les expertises ordonnées par les conseils de prud'hommes et par les juridictions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Tout à fait ! Cet article ne fait donc que mettre en oeuvre, pour les expertises ordonnées par les tribunaux de grande instance et par les cours d'appel, le monopole dont la CDC bénéficie déjà en application d'une ordonnance de 1816. L'accomplissement de cette tâche ne nécessitant aucun accueil des justiciables, l'accès au service public de la justice ne sera pas entravé. Les justiciables bénéficieront toujours, en outre, de l'accueil physique proposé dans les juridictions, qui conserveront l'intégralité de leur dossier et pourront utilement les renseigner. Le transfert à la Caisse des dépôts de ces tâches, qui sont réalisées manuellement dans les greffes, sera source d'importants gains de temps pour les greffiers, lesquels pourront ainsi consacrer plus de temps à leurs autres attributions au bénéfice des justiciables. Des échanges sont en cours entre la Caisse des dépôts et le ministère de la justice pour affiner le projet. C'est un travail qui mérite d'être mené et qui rendra nos juridictions plus efficaces.

à la Caisse des dépôts la gestion de certaines saisies sur rémunération, ainsi que des sommes consignées pour expertise. La commission a souhaité supprimer cet article 9. Le transfert est uniquement justifié pour des raisons de charge de travail, les greffes en charge de ces missions ne pouvant plus les assumer de façon satisfaisante. C'est notamment le cas pour les procédures impliquant une régie d'avances et de recettes. Si nous comprenons les dysfonctionnements qui peuvent exister, la solution proposée ne nous paraît,

En outre, la légitimité de la CDC à répartir les saisies sur rémunération ne nous paraît pas certaine. Nous avons donc émis un avis quelque peu défavorable, dirai-je.

de simplifier la procédure d'expulsion s'agissant du sort des meubles de la personne expulsée. La procédure de saisie immobilière a été profondément réformée en 2006. Il est aujourd'hui temps d'ajuster certaines de ses dispositions pour améliorer son fonctionnement. Une large consultation a été menée à ce sujet avec le barreau, des magistrats, des greffiers et des professeurs de droit. L'amendement que je vous présente en est le fruit. Il vise à organiser la saisie simultanée de plusieurs immeubles du débiteur par un même créancier et à faciliter l'établissement du titre de vente par le notaire en cas de vente amiable. la vente de gré à gré est désormais autorisée après le jugement d'orientation, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Actuellement, lorsque le débiteur n'a pas réussi à vendre son bien à l'amiable dans le délai fixé par le juge, la vente sur adjudication de l'immeuble est ordonnée. Or sa vente aux enchères occasionne des frais qui sont à la charge du débiteur, et qui aggravent sa situation financière. Les frais de publicité peuvent ainsi parfois dépasser la somme de 10 000 euros. En outre, le prix de vente à la barre est parfois décevant, en raison du faible nombre d'enchérisseurs. Pourtant, il arrive que le débiteur trouve un acquéreur entre le jugement ordonnant son adjudication et l'ouverture des enchères. L'autoriser à vendre son bien de gré à gré, avec l'accord de ses créanciers, permettra ainsi de vendre le bien à un meilleur prix au bénéfice de l'ensemble des parties. En matière d'expulsion, le juge statue systématiquement sur le sort des biens de la personne expulsée après une audience. En l'absence de contestation de la personne expulsée, le juge ne peut qu'ordonner la vente aux enchères publiques des biens qui ont une valeur marchande, et déclarer abandonnés les autres biens sur la base de l'inventaire réalisé par l'huissier de justice dans le procès-verbal d'expulsion. L'intervention du juge de l'exécution n'apporte, dans ce cas, pas de plus-value, mais elle engendre des frais. L'audience ne sera donc maintenue qu'en cas de contestation. Nous proposons donc en réalité une amélioration sensible de cette procédure au bénéfice des justiciables, en premier lieu de ceux qui, déjà en situation difficile, sont confrontés à une saisie de leurs biens immobiliers.

La requête en divorce est supprimée pour unifier le régime procédural. En effet, il ne nous semble pas utile de distinguer deux phases : la phase de conciliation sur les mesures provisoires et celle qui suit au fond. La réduction de la durée de la procédure qui en découlera nécessairement est un souhait constant des justiciables, qui déplorent régulièrement la durée excessive des procédures judiciaires en divorce. Cette durée est aujourd'hui estimée à peu près à trente mois ; elle devrait être divisée par deux grâce à la procédure que je vous propose. Pour les greffes, il en résultera une simplification du travail de gestion des dossiers et de la saisie informatique. Ce temps gagné sur un travail purement administratif sera du temps consacré à l'accueil, à l'écoute des personnes et à la préparation des dossiers. En outre, cette réforme s'inscrit dans le cadre des évolutions réelles de la société. Le rôle du juge n'est plus aujourd'hui de tenter une conciliation sur le principe même du divorce, en se penchant sur les raisons du démariage ou de la séparation des couples. Le juge doit, en revanche, se consacrer aux conséquences juridiques des situations qui sont vécues par ces couples et des décisions qu'ils souhaitent prendre. Dans ce contexte, je tiens à l'affirmer avec force, les mesures provisoires et l'accès au juge sont préservés. Toutes les mesures qui peuvent être aujourd'hui prononcées lors de l'ordonnance de non-conciliation pourront l'être dans le nouveau cadre procédural, après la saisine du juge aux affaires familiales. Cela aura lieu lors d'une audience sur les mesures provisoires, qui sera tenue à la demande d'au moins l'une des deux parties. Je le dis clairement, la présence des parties à l'audience sera possible et pourra aussi être ordonnée par le juge. Dans ce nouveau cadre procédural, le rôle assigné au juge pour concilier les parties sur les décisions provisoires utiles et nécessaires permettra de s'assurer du respect de l'intérêt des enfants et de veiller à l'équilibre entre les intérêts des époux. Tout cela, bien entendu, est maintenu. Par ailleurs, il faut continuer à inciter les parties à recourir à des divorces moins conflictuels, dans l'esprit de la réforme du divorce de 2004. Nous proposons donc que la demande en divorce n'en mentionne pas la cause, sauf lorsqu'il s'agit d'un divorce accepté ou lié à une rupture ancienne. Le fondement du divorce, c'est-à-dire sa cause, ne sera indiqué, au plus tôt, qu'au moment des premières écritures au fond. Vous le constatez, cette réforme répond aux impératifs de simplification procédurale que je souhaite réellement porter, tout en préservant les avancées d'apaisement qui découlent de la loi de 2004. Cette proposition de réforme consacre le rôle du juge du divorce dans ses missions tant d'écoute des personnes que d'encadrement juridique des séparations. Elle permettra de gagner du temps, tout en respectant les parties concernées.

la disposition que vient de défendre Mme la ministre, et qui tend à l'allégement de la procédure de divorce contentieux par la suppression du préalable obligatoire de la conciliation. Cet amendement participe de la volonté de simplification et d'unification de l'instance civile. Cette disposition est particulièrement opportune dans un contexte qui voit émerger le nouveau divorce par consentement mutuel, lequel se déroule désormais, hors quelques hypothèses il existe une demande d'audition d'enfant, en dehors du cadre judiciaire. Il convient en effet de moderniser le cadre procédural des divorces contentieux afin d'améliorer la lisibilité de la procédure et de réduire les délais de traitement. Il ne fait guère de doute que la suppression de la tentative de conciliation accélérera la procédure et contribuera à désengorger les tribunaux. Cette suppression sera compensée par la possibilité d'obtenir du juge

La mission interministérielle pour la protection des femmes contre la violence et la lutte contre la traite des êtres humains souligne régulièrement l'importance du phénomène. Pour l'année 2016, elle a ainsi relevé que 123 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint quatre cinquièmes des victimes de violences ne déposaient pas de plainte, ce qui porterait leur nombre à près de 500 000 personnes, hommes et femmes. Les instruments juridiques existants doivent être améliorés. On peut facilement imaginer que les victimes de violences conjugales soient plus particulièrement exposées pendant les séparations ou que ces violences se déclenchent au moment de la demande d'un divorce. Ainsi, les victimes de violences conjugales peuvent être tentées d'accepter un divorce par consentement mutuel devant notaire par volonté de se prémunir contre ces violences, sans qu'un juge puisse prononcer des mesures provisoires qui les protégeraient. également probable que l'accord obtenu par la convention leur soit moins favorable qu'une décision de divorce pour faute. Dans cette perspective, nous proposons de réfléchir à un mécanisme qui pourrait permettre d'alerter un juge de l'existence de telles violences au cours d'un divorce par consentement mutuel, sans risquer d'exposer les victimes à d'éventuelles représailles. Quel

Finalement, à un problème de temps de procédure, c'est-à-dire de durée de convocation à une audience de conciliation, on apporte une solution simple,

puisqu'il prévoit que le notaire, informé par l'avocat de l'un des époux de violences au sein d'un couple qui divorce par consentement mutuel, saisirait le juge aux affaires familiales en urgence. Ce n'est évidemment pas le rôle du notaire ! L'avocat

d'une intention tout à fait louable, il me semble méconnaître le dispositif du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire. L'un des apports majeurs de cette réforme, qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2017, est d'avoir prévu que chacun des doit avoir son propre avocat pour bénéficier d'un conseil personnalisé et indépendant. L'obligation ainsi créée équilibre vraiment ce nouveau divorce.

Cet auxiliaire de justice pourra aussi l'accompagner pour une saisine urgente du juge aux affaires familiales selon la procédure dédiée de l'ordonnance de protection, qui est extrêmement utile, ce qui sera en outre beaucoup plus efficace et rapide qu'une transmission de saisine par le notaire. De plus, le notaire, officier public et ministériel, vous le savez, est tenu par l'article 40 du code de procédure pénale d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a connaissance.

de vote. Sur ce point, madame la ministre, je crois quand même qu'il y a une ambiguïté. En effet, depuis que nous avons entamé l'examen de ce texte, on nous a beaucoup parlé de conciliation,

ne m'explique pas. Supprimer la conciliation, alors que nous sommes dans un domaine où l'on doit à tout prix la rechercher, ne serait-ce que dans l'intérêt des enfants, est complètement contradictoire avec ce qu'on nous a dit depuis le début du débat sur la médiation

Le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel a suscité- et suscite encore - des craintes ou, du moins, des interrogations chez les juristes et praticiens du droit

À mon sens, il serait nécessaire- utile, en tout état de cause -, mais surtout urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce

1° et 2° du paragraphe I, qui ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant, bien entendu, toute action en nullité susceptible de la remettre en cause pour ce qui est des conséquences attachées au divorce. L'amendement

En l'absence d'une intervention du juge, il est désormais susceptible d'être remis en cause, notamment par le biais d'une action en nullité de droit commun pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d'un notaire. Mes chers collègues, ans pour des gens qui ont le sentiment d'être divorcés parce qu'ils ont décidé de le faire, vous conviendrez que c'est long Pendant ce délai, les époux divorcés par consentement mutuel conventionnel- divorce, je le répète, non homologué par un juge -peuvent se remarier. Pendant cinq ans, ils peuvent refaire des enfants. Afin de ne pas troubler ce que j'appelle « l'aura pacifique escomptée », il me paraît nécessaire de sécuriser ce divorce en réduisant le délai de prescription de l'action en nullité

d'encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l'égard de leurs enfants de manière négociée et discutée- et ce, toujours pour simplifier en amont de toute intervention judiciaire -, cet amendement vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d'un notaire

conciliateur et à permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l'égard de leurs enfants avant d'envisager,

créée par les dispositions de la loi de 2016, dite loi de modernisation de la justice du XXI siècle. Sur l'opportunité des modifications proposées, nous tenons à souligner que, si des critiques ont pu s'élever concernant le principe de la déjudiciarisation de ce mode de divorce

Si le dépôt confère date certaine et force exécutoire à la convention, le notaire ne fait que constater le divorce. Il ne le prononce pas, comme le faisait le juge. C'est bien l'accord des époux, inscrit dans la convention, qui réalise le divorce.

des vérifications auxquelles sont tenus les avocats, puisque les majeurs sous mesure de protection ne peuvent pas recourir au divorce par consentement mutuel sans juge. Les avocats, dès lors qu'ils agissent au nom et pour le compte de leurs clients, peuvent, au même titre que les notaires, avoir accès aux copies intégrales d'actes d'état civil de ces derniers. Cette demande peut même être dématérialisée. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement à l'amendement n° 6 rectifié, qui concerne le délai de prescription d'un an des actions en nullité dirigées contre les conventions de divorce par consentement mutuel que nous venons d'évoquer. En application du droit commun, ce délai est aujourd'hui de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir. Les auteurs de l'amendement proposent donc un changement considérable de nos règles de prescription. Or nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que ce changement préserverait l'équilibre entre les différents intérêts à protéger. Ne risque-t-on pas- la commission s'est d'ailleurs posé la question -d'avoir un divorce judiciaire très protecteur des intérêts des parties- notamment des parties les plus faibles -grâce au contrôle du juge et, inversement, d'avoir un divorce par consentement mutuel très peu protecteur, puisque sans contrôle du magistrat et attaquable seulement dans un délai d'un an

déjudiciarisé, c'est-à-dire le recours à cet acte sous seing privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, aux décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés. Cette extension est très importante, puisque l'ensemble de ces mesures seraient alors, elles aussi, soustraites

par M. le rapporteur et que je partage globalement. Je voudrais simplement dire ici que les évolutions que vous proposez relatives au divorce par consentement mutuel sans juge forment un

il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu'à une simple séparation de corps. Cet amendement vise donc,

Les points 1° à 6° de cet amendement visent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Qui peut le plus peut le moins

duquel « en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel ». On enferme ainsi les époux. Supposez qu'il

Cet amendement vise à ouvrir une exception à ce principe s'agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298

par consentement mutuel et non pas les divorces judiciaires. La convention qui les acte doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble. Ce rendez-vous commun, où chacun est présent, me semble fondamental pour s'assurer du consentement de tous, au même moment, à l'intégralité des dispositions de la convention. Le recours à la signature électronique me semble-t-il, que le divorce intervienne sans que les parties se rencontrent, alors qu'il s'agit d'un consentement mutuel que nous cherchons à acter. En outre, la présence des époux permet aux avocats de s'assurer de l'identité des signataires, ce qui est indispensable s'agissant d'un acte qui touche à l'état des personnes. Pour toutes ces raisons, le recours à l'acte électronique en matière familiale me paraît peu souhaitable. Je reste attachée à ce que, en cette matière qui touche à l'intime des familles, le progrès numérique ne conduise pas à une forme de déshumanisation des séparations.

exprès des parties, se dérouler sans audience, et donc exclusivement par voie écrite. Corrélée au sort réservé au tribunal d'instance par le projet de loi organique, cette disposition vise l'ensemble des procédures, quel que soit le montant impacté. Cela porte gravement atteinte au principe de l'oralité des débats, qui pourraient, pour des raisons « pratiques », progressivement disparaître. L'argument principal souvent invoqué pour justifier ce passage à une procédure exclusivement écrite est la contrainte que représenterait la compétence territoriale- contrainte pour les parties. Or cet argument se heurte à deux impasses. Tout d'abord, la mise en place du service d'accueil unique du justiciable, le SAUJ, et l'extension de son périmètre d'intervention à l'ensemble du territoire national devraient permettre de déposer la requête dans n'importe quel tribunal, à charge pour l'institution de la transmettre à la juridiction territorialement Il serait donc opportun d'attendre la mise en place de ce dispositif et d'en mesurer ses effets. Ensuite, l'importance de l'audience est négligée : pour reformuler les demandes des parties, tenter de les concilier et aboutir à une solution judiciairement acceptée, le cadre de la procédure orale est parfaitement adapté et son maintien paraît plus que souhaitable. Par ailleurs, ce même article prévoit que les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini en Conseil d'État peuvent, avec l'accord des parties, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience. Aux termes le tribunal pourra toutefois décider de tenir une audience si les preuves écrites ne sont pas suffisantes ou à la demande des parties. Mais s'il estime qu'une audience n'est pas nécessaire, le tribunal pourra rejeter la demande d'audience d'une des parties par décision spécialement motivée. Ces dispositions sont contestables, qu'il s'agisse de l'instauration d'une saisine et d'une procédure intégralement dématérialisées pour les parties ou de la disparition

montant. Nous avons apporté des garanties en commission, notamment la possibilité pour les parties de revenir à la procédure ordinaire si elles estiment finalement que le dossier soulève des difficultés. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable

je le rappelle, devront y consentir expressément. Cela sera possible dans deux hypothèses distinctes. De manière générale, De manière générale, devant le tribunal de grande instance, les parties pourront renoncer à l'audience. Je rappelle que tel est déjà le cas lorsque, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire, les avocats remettent leur dossier au tribunal. C'est également possible lorsque, devant le le juge autorise les parties qui ont comparu à une audience précédente à ne pas se présenter de nouveau. Le projet de loi tend donc à généraliser une telle possibilité, si les parties le souhaitent. Par ailleurs, les parties qui ont recours à la procédure dématérialisée de traitement des petits litiges accepteront de se placer dans une procédure sans audience. Pour ces

pour procéder à l'audition des parties ou à une vérification d'écriture, ou bien si une partie en fait la demande. Dans ce dernier cas, le juge a le pouvoir de refuser la tenue d'une audience qui lui paraîtrait inutile, mais cette décision, spécialement motivée, sera susceptible de recours. Les principes fondamentaux du procès sont donc respectés.

en fait explicitement la demande, il tient une audience.

Nous considérons que l'audience possède non pas uniquement une utilité procédurale, mais également une utilité sociale, puisque le justiciable y obtient la résolution d'un litige par un juge représentant la République. Pour de nombreux justiciables, le sentiment d'avoir été entendus contribue au sentiment de justice, y compris lorsque la décision finale leur est défavorable. L'audience peut permettre aux magistrats de préparer le requérant à leur décision. C'est pourquoi nous considérons qu'il serait malvenu de raisonner à partir d'un seuil objectif pour déterminer le champ de la procédure écrite en la matière. Il serait

Cet amendement vise à substituer la mention du seuil défini par décret en Conseil d'État, par celle d'une « créance dont l'existence ou l'ordre de grandeur n'est pas contestée par l'une des parties

cet amendement, il s'agit de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, de refuser de tenir une audience. La commission des lois a complété l'article 13 du projet de loi, en précisant que, devant le tribunal de grande instance, le juge devait conserver la possibilité de tenir une audience alors que les parties étaient expressément d'accord pour pour que la procédure se déroule sans audience. Il convient en effet de préserver ce pouvoir du juge, gardien du procès équitable. Toutefois, dans la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité pour le tribunal de refuser de tenir une audience, lorsque cette demande émane de l'une des parties et que le juge estime que celle-ci n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

Il prévoyait qu'elle s'appliquerait à tous les litiges civils inférieurs à 4 000 euros, qu'il s'agisse des conflits de voisinage, de la consommation, d'injonctions de payer ou de faire, et qu'une décision judiciaire serait rendue dans les deux mois, à défaut de conciliation. Cette proposition du Président de la République figure également également dans le rapport issu des chantiers de la justice consacré à la procédure civile, que m'ont rendu Mme Agostini et M. le professeur Molfessis, pour l'amélioration et la simplification de la procédure civile. L'objectif poursuivi est également de transposer en droit interne une procédure issue d'un règlement européen instituant une procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers. Il s'agit d'un règlement de 2007, modifié le 16 décembre 2015. Les justiciables pourront ainsi obtenir une décision dans un délai raccourci, grâce à des échanges s'effectuant de manière complètement dématérialisée le portail de la justice. Je tiens ici à vous rassurer, il ne s'agit pas de tenir les parties à distance du juge : la procédure dématérialisée pourra constituer un véritable progrès

notamment au vu des pièces produites par son adversaire. Toutefois, on peut imaginer des hypothèses où l'audience sera manifestement inutile ou bien s'analysera en une demande dilatoire, à l'issue de la procédure dématérialisée. Enfin, le refus du juge de tenir une audience pourra, avec la décision rendue au fond, faire l'objet d'un recours. Je crois qu'il faut faire confiance au juge. Gageons qu'il ne refusera pas une audience. S'il le fait, c'est que celle-ci lui apparaîtra manifestement inutile. Quel